La séance est reprise. J'ai reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République en date du 18 juin 2018 portant convocation du Parlement en session extraordinaire à compter du 3 juillet 2018. Le décret vous a été communiqué. La conférence des présidents, qui se réunira demain à dix-neuf heures trente, établira le programme de la session extraordinaire. communication. J'ai reçu de M. le Président de la République une lettre m'informant de sa décision de s'adresser, en application du deuxième alinéa de l'article 18 de la Constitution, aux membres du Parlement réunis à cet effet en Congrès le lundi 9 juillet

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie

Le contexte politique sur notre continent étant actuellement très instable, pour ne pas dire critique- le risque pour l'Union européenne est de se disloquer autour de la question des migrations -, vous comprendrez que la présence de Gérard Collomb à cette réunion de haute importance

mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie qui vous est soumis est donc un texte très important. très important, car il s'agit de permettre à toutes celles et à tous ceux qui fuient la guerre et la persécution d'être mieux accueillis en France, de voir leurs démarches facilitées et de commencer plus tôt leur parcours pour s'insérer dans la société française. très important, car les mesures que nous allons examiner visent aussi à lutter contre l'immigration illégale, ce qui correspond, vous le mesurez dans vos territoires, à une aspiration forte exprimée par nos concitoyens, aspiration à laquelle nous devons répondre si nous ne voulons pas que, demain, tous les populismes grandissent encore dans notre pays. C'est vrai ! Sur ces questions sensibles, je crois que nous serons tous d'accord, au sein de la Haute Assemblée, pour souligner qu'on ne saurait se soumettre au diktat de l'image et de la peur. Oui, pour penser des solutions pertinentes au défi migratoire, il convient de se fonder sur une analyse objective de la situation.

en 2015 et de 1,2 million en 2016, ont diminué de moitié l'année dernière pour s'établir à 600 000. Les franchissements illégaux des frontières extérieures de l'espace Schengen s'établissent, eux, à un niveau certes élevé-

Toutefois, il convient de demeurer vigilant, car on constate depuis quelques mois une forte recrudescence des flux migratoires sur la route orientale et sur la route occidentale. un épisode comme celui que nous avons vécu la semaine dernière avec l'a révélé que la route migratoire de Méditerranée centrale, si elle est moins empruntée qu'auparavant, demeure très active. La crise migratoire en Europe est donc loin d'être terminée. En France, la situation est encore plus préoccupante, car on observe une évolution à contre-courant de celle que je viens de décrire.

Notre territoire est de plus en plus exposé à des flux secondaires de dizaines de milliers de personnes qui, s'étant vu refuser l'asile dans un autre pays européen, viennent tenter leur chance sur notre sol. Les conséquences de cette situation, vous les vivez au quotidien dans vos territoires. Notre dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile est saturé, alors même que le nombre de places disponibles a doublé en quelques années, passant de 44 000 en 2012 à 80 000 aujourd'hui.

au coeur de nos villes, grandes et moyennes, se multiplient des campements de fortune où, pour les migrants, les conditions de vie sont très difficiles, et qui, pour les riverains, sont hélas générateurs d'importantes nuisances, voire de troubles à l'ordre public,

constat objectif. Agir, c'est ce que le Président de la République et le Gouvernement ont fait depuis un an en travaillant en Afrique, auprès des pays d'origine des migrations. République a ainsi pris des initiatives fortes pour contribuer à stabiliser le continent africain et pour éviter que n'y naissent de nouveaux conflits qui seraient nécessairement porteurs de nouvelles migrations. La France et l'Union européenne s'engagent pour donner un avenir à la jeunesse africaine, notamment au travers de l'aide au développement- telle était la teneur du discours du Président de la République à Ouagadougou. Nous sommes également en pointe pour lutter contre les réseaux de passeurs. Il ne faut pas croire en effet que les migrations sont exclusivement des mouvements spontanés. Elles sont aussi le fruit de l'action de trafiquants d'êtres humains, souvent liés au crime, au commerce des armes, voire au terrorisme, qui dépouillent les migrants de tous leurs biens, les font passer par des routes dangereuses au coeur du désert, les placent dans des camps en Libye, avant de leur faire tenter une traversée plus que périlleuse de la Méditerranée. Contre cela, oui, nous nous devons de lutter, et nous luttons. La France est par ailleurs très active aux portes de l'Union européenne, grâce à l'action résolue conduite par le ministre d'État, ministre de l'intérieur, pour faire en sorte que les ressortissants de pays comme l'Albanie qui bénéficient d'une exemption de visa ne détournent pas cette facilité pour demander l'asile en Europe, alors même que leur taux de protection est extrêmement faible, aux alentours de 5 %. Nous avons obtenu de premiers résultats puisque la demande albanaise a baissé d'un tiers entre les premiers mois de 2017 et les premiers mois de 2018. Enfin, nous travaillons aussi avec nos partenaires européens, même si le récent contexte politique complexifie notre action, notre action, afin que se développe une véritable solidarité européenne en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Il convient donc, mesdames, messieurs les sénateurs, d'agir à l'échelon international, car la réponse au défi migratoire est et sera nécessairement globale. Mais si la France est aujourd'hui à contre-courant des autres nations européennes, avec une demande en hausse quand celle-ci baisse partout ailleurs, c'est parce que notre système d'asile et d'immigration est perfectible. Depuis un an, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures fortes pour améliorer ce dernier. Je rappelle que le renforcement des moyens des services des étrangers des préfectures, la création dans chaque grande région de centres d'accueil et d'examen des situations, les CAES,

Lors de la campagne présidentielle, le Président de la République avait pris l'engagement fort de réduire à six mois en moyenne le délai d'instruction de la demande d'asile. Il voulait, soulignait-il, permettre à ceux qui obtiendront une protection de commencer rapidement leur parcours d'intégration dans la société française

projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie a fait l'objet d'une large adoption par les députés le 22 avril dernier. À l'issue de débats qui se sont tenus pendant près d'une semaine, les députés sont parvenus à l'adoption d'un texte que nous considérons comme équilibré. Le projet de loi a ensuite été largement amendé lors de son examen le 6 juin par la commission des lois le rapporteur, François-Noël Buffet. Certains enrichissements vont dans le bon sens, et le Gouvernement proposera qu'ils soient conservés. Il est en revanche des mesures qui, de nature à remettre en cause l'équilibre du texte entre humanité et efficacité, recevront de notre part un avis défavorable. Sur les points les plus symboliques, le Gouvernement a déposé des amendements qui tendent soit à revenir à l'esprit du texte initial, soit à supprimer certaines dispositions avec lesquelles il ne peut être en accord.

les dispositions portant d'un à quatre ans la durée de validité des titres de séjour délivrés aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides et revenir sur la possibilité pour les frères et les soeurs d'un réfugié mineur- je parle bien d'un réfugié reconnu comme tel au titre de l'asile -de le rejoindre.

qu'il ne faut pas confondre ce public avec les mineurs non accompagnés, pris en charge par les conseils départementaux au titre de l'aide sociale à l'enfance. La portée de cette disposition ne doit donc pas être surestimée. Le Gouvernement ne peut évidemment accepter sa suppression, car c'est la grandeur de la France que de proposer de telles mesures, qui ciblent les personnes les plus vulnérables et sont conformes à la grande tradition d'accueil de notre pays. ensuite des mesures dont la portée opérationnelle ne me semble absolument pas garantie et qui emportent plus d'inconvénients juridiques que d'avantages.

me semble entraîner une certaine confusion entre, d'une part, la portée de la décision prise par l'OFPRA ou la CNDA et, d'autre part, les prérogatives de l'autorité administrative. ! J'ai également à l'esprit l'instauration de quotas, qui ne furent pas mis en oeuvre sous de précédentes législatures, alors même que les occasions n'auraient pas pas manqué de le faire lors des nombreuses modifications du droit des étrangers dont le Parlement avait été saisi. Comment le Gouvernement pourrait-il accepter une telle évolution ? ? La limitation du droit au regroupement familial que la mise en place de quotas occasionnerait est directement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier à son article 8, qui reconnaît le droit à une vie familiale normale. De même, vous proposez de supprimer l'aide médicale de l'État et de la remplacer par une aide médicale d'urgence, dont le panier de soins serait plus réduit. également, le Gouvernement ne saurait admettre une telle régression des droits des personnes qui aurait pour conséquence, en réduisant les soins accordés aux étrangers, fussent-ils en situation irrégulière, d'accroître les risques pour la santé publique en général.

Mesdames, messieurs les sénateurs, l'enjeu qui nous réunit aujourd'hui est tout à fait décisif pour la France et pour les Français, bien sûr, pour lesquels la question migratoire est une des préoccupations principales, mais, plus largement, pour l'avenir de l'Europe. On voit quelles positions sont en présence. Il y a d'abord ceux qui souhaitent accueillir tous ceux qui veulent venir et nient jusqu'à l'existence même des frontières. C'est là, chacun le comprend, une impasse, car l'Europe ne pourra jamais faire face, par exemple, au doublement de la population de l'Afrique. Il y a ensuite ceux- ils sont de plus en plus nombreux en Europe et en France -qui rejettent tout accueil, y compris celui de personnes qui fuient la guerre et la persécution. Cela est en tout point contraire à l'histoire européenne et jamais nous n'accepterons que le droit d'asile soit remis en question. La responsabilité de la France est de porter une ligne empreinte de fermeté et de justice, d'efficacité et d'humanité, fidèle aux valeurs de la République, fidèle aux valeurs de l'Europe, qui en a besoin.

qui est présenté devant le Parlement sur cette thématique, dont seize projets de loi majeurs, les derniers datant de 2015 et de 2016.

au député Aurélien Taché. Sur le fond, les enjeux européens et internationaux des politiques migratoires sont totalement ignorés. Aucune mesure n'est prévue pour faire pression sur certains de nos partenaires, notamment pour l'obtention de laissez-passer consulaires ou pour encourager la participation de la France au mécanisme de solidarité européen.

De même, ni le Gouvernement ni les parlementaires de la majorité à l'Assemblée nationale n'ont eu le courage de traiter la situation des mineurs placés en centre de rétention avec leur famille, ouvrant même la possibilité de les retenir trois mois, dans des lieux totalement inadaptés. L'intégration est donc le parent pauvre de ce texte. La formation linguistique à destination des étrangers en situation régulière est en moyenne de 148 heures, contre 242 heures en 2012. Même si le Gouvernement doublait le nombre d'heures de français, nous serions très loin de l'Allemagne, qui dispense 600 heures de formation linguistique aux étrangers primo-arrivants et jusqu'à 900 heures aux réfugiés.

Je ne saurais continuer sans rappeler le contexte dans lequel nous nous trouvons. L'Europe a connu depuis 2015 une vague d'arrivées sur son territoire d'une ampleur inédite depuis la Seconde Guerre mondiale et le conflit de l'ex-Yougoslavie

l'Union européenne et la Turquie du 18 mars 2016, à la mise en place de et au programme temporaire de relocalisation destiné à soulager l'Italie et la Grèce. À l'échelle de l'Europe, la demande de protection internationale subit une baisse comparable et s'est établie en 2017 à 706 000 demandes d'asile, une diminution de 43 % par rapport à 2016. Cette évolution numérique s'accompagne d'une reconfiguration géographique des principales routes de migration vers l'Europe. Les flux en Méditerranée centrale ont connu une diminution notable- moins 32 % entre 2016 et 2017. Il en va de même en Méditerranée orientale. En revanche, le flux passant par la Méditerranée occidentale est en nette augmentation. Fortement exposée par sa situation géographique aux flux dits « secondaires » ou « de rebond » internes à l'Union européenne, la France connaît désormais une demande d'asile à la hausse, alors même que celle-ci tend à se stabiliser chez ses voisins : 100 412 demandes en 2017, soit une augmentation de 17,1 % depuis 2016. De même, la délivrance de premiers titres de séjour a connu une hausse ininterrompue depuis 2012, particulièrement forte en 2016 et en 2017.

En matière d'éloignement, nos systèmes sont en surchauffe et nos dispositifs sont sursollicités : le taux d'occupation des centres de rétention s'établit cette année à 81 % et s'accompagne d'une gestion des escortes et des transferts à flux tendus.

au Parlement chaque année ; de resserrer les conditions du regroupement familial ; de transformer- oui ! -l'aide médicale de l'État en aide médicale d'urgence et de mieux identifier les secteurs économiques en manque de main-d'oeuvre.

une immigration régulière et traiter les demandes d'asile dans de bonnes conditions, au profit de ceux qui doivent en bénéficier, si l'on n'est pas capable de tenir un discours ferme à l'encontre de ceux qui entrent irrégulièrement sur le territoire et qui entendent y rester. C'est la raison pour laquelle

refusé d'affaiblir le délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier sur le territoire, ainsi que cela avait été fait à l'Assemblée nationale. S'agissant des mineurs étrangers, nous interdisons explicitement le placement en rétention de mineurs isolés

l'initiative de sa présidente, Mme Catherine Morin-Desailly, le bureau de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a décidé de rendre un avis sur ce texte transmis au fond à la commission des lois, mais dont quelques dispositions intéressent tout particulièrement notre commission, dans ses compétences relatives à l'éducation, à la jeunesse, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la culture.

l'article 21, relatif à la mobilité des étudiants étrangers et à l'autorisation provisoire de séjour qui leur permet aujourd'hui de rester douze mois supplémentaires sur le territoire après l'obtention de leur diplôme pour chercher un emploi ou créer une entreprise,

En 2015, lors de nos travaux sur le projet de loi relatif au droit des étrangers en France, la commission de la culture avait marqué son attachement aux dispositifs d'immigration choisie, lesquels permettent d'attirer en France des talents étrangers qui contribuent ensuite à faire rayonner notre pays à l'international. La France peut s'enorgueillir d'accueillir plus de 73 000 étudiants étrangers chaque année, ce qui la place au quatrième rang mondial et au premier rang des pays non anglophones.

C'est un véritable risque, madame le ministre, et des mesures doivent être prises pour garantir un codéveloppement des talents internationaux. Permettez-moi enfin d'attirer votre attention sur le fait que le développement des dispositifs d'immigration légale choisie doit se faire avec rigueur. En ces temps de pression migratoire forte sur les pays de l'Union européenne, les risques de détournement des dispositifs doivent être bien appréciés, et l'immigration légale doit être également contenue. Il y a bientôt trois semaines, la commission de la culture a examiné le projet de loi et adopté huit amendements, qui ont tous été intégrés dans le texte de la commission des lois que nous examinons aujourd'hui.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la migration est un phénomène aussi ancien que l'humanité. Nous n'empêcherons pas les femmes et les hommes de migrer, d'autant moins que les conflits internationaux, l'ordre économique libéral établi et les bouleversements climatiques font de notre monde un monde de réfugiés. Renforcer les opérations de police aux frontières et la politique d'expulsion ne changera rien à cet état de fait. Ces femmes et ces hommes qui migrent ne le font sûrement pas pour bénéficier de telle ou telle aide sociale, qu'ils compareraient selon les pays. Madame la ministre, lorsque l'on essaie de fuir la violence, la torture, la guerre, la famine, les catastrophes écologiques, quitter son pays, ses amis, et sa famille parfois, représente une vraie souffrance. rien ne décourage ces femmes et ces hommes qui cherchent simplement à vivre ailleurs, car ils y sont contraints, rien, pas même la violence des frontières qui se ferment devant eux. La fonte des neiges dans les Alpes nous l'a récemment rappelé, en révélant les dépouilles de corps de migrants contraints d'emprunter des détours en pleine montagne ; ces mêmes migrants que certains extrémistes nationalistes chassaient fièrement à bord d'hélicoptères il y a peu ; ces mêmes que d'autres citoyens, plus fidèles aux valeurs de notre République, aident en toute fraternité, avant d'être traînés devant les tribunaux ! Votre conception de la politique migratoire s'inscrit dans un projet plus global vous vous attaquez à la solidarité des Français envers les étrangers comme vous montez les Français les uns contre les autres, pour servir les intérêts d'une politique de libéralisation et de casse des valeurs républicaines, droit d'asile compris. L'attitude de la France et de l'Europe met en danger les migrants et laisse les citoyens et les associations gérer l'urgence humanitaire. C'est ainsi que ces 629 femmes et hommes rescapés, repêchés en mer par l', n'ont trouvé d'accueil ni en Italie ni en France 629 femmes et hommes qui « ne sont rien » et qui méritent sans doute d'être « responsabilisés », mis au pas, comme le sont les Français sous le régime de La République En Marche.

l'heure n'est pas à l'apaisement, comme l'a déclaré Emmanuel Macron, puisque, juste après sa rencontre avec le chef du gouvernement italien, Rome refusait une nouvelle fois l'accès de ses ports à des bateaux d'ONG. Aujourd'hui, madame la ministre, l'émotion et la colère sont d'autant plus fortes et légitimes que votre texte enfreint un certain nombre de principes fondamentaux, à commencer par le droit d'asile, qui fait partie intégrante de l'histoire démocratique française. La Constitution du 24 juin 1793 proclamait déjà que le peuple français « donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. -Il le refuse aux tyrans. l'acte fondateur du droit d'asile, élément constitutif des grands principes de la Révolution française et du siècle des Lumières. Quel tralala ! Faut-il rappeler ces mots de Voltaire dans son ? « Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères ! Le droit d'asile est désormais consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, forgée par la Résistance : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. C'est en se fondant sur ce texte que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 août 1993, a qualifié le droit d'asile d'« exigence constitutionnelle ». Peu après cette décision, la révision constitutionnelle du 25 novembre 1993, nécessaire à la pleine application par la France de la convention de Schengen, a inscrit dans la Constitution un article 53-1 aux termes duquel les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Loin des faux bons sentiments, la logique de pénalisation et de sanction des demandeurs d'asile que développe ce projet de loi enfreint cette tradition d'asile du droit français. Il est porté atteinte au droit d'asile dans la phase administrative de la demande comme dans sa phase contentieuse. Premièrement, le texte, en son article 5, entrave le dépôt de la demande d'asile dans un délai raisonnable et ne permet pas la bonne information des demandeurs d'asile quant au sort qui leur est réservé. Deuxièmement, l'article 6 porte gravement atteinte au droit au recours effectif des demandeurs d'asile en réduisant le délai pour exercer un recours devant la CNDA, le Gouvernement souhaitant rétablir par voie d'amendement la réduction, supprimée par la commission des lois, Cette réduction excessive des délais conduit à une justice expéditive. Pourtant, le 2 février 2012, la Cour européenne des droits de l'homme rendait un arrêt de condamnation à l'encontre de la France, considérant que la procédure prioritaire alors prévue pour l'examen de certaines demandes d'asile n'était pas conforme au droit au recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Troisièmement, l'article 8 du présent projet de loi met fin au caractère suspensif de certains recours devant la CNDA. Celui-ci était pourtant consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993 : « Considérant que le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d'une manière générale que l'étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. » Quatrièmement, sera possible d'imposer au demandeur d'asile tout au long de la procédure une langue qui n'est pas la sienne, sans que soient respectés ni les garanties procédurales européennes ni le droit de tout justiciable à être entendu dans une langue maîtrisée. Cinquièmement, en plus d'entraver davantage la procédure d'examen de la demande avec la fin de la notification des convocations et décisions par lettre recommandée, le texte prévoyant que cette notification faire « par tout moyen », le Gouvernement ne respecte pas le principe de confidentialité que le Conseil constitutionnel a érigé au rang de « garantie essentielle du droit d'asile », principe de valeur constitutionnelle. Sixièmement, le projet de loi supprime le caractère facultatif de la visioconférence en l'imposant aux justiciables. Une telle généralisation est encore une fois parfaitement contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Saisis notamment de la question du recours à la visioconférence pour les audiences de prolongation de rétention administrative, les sages ont jugé, dans une décision du 20 novembre 2003, qu'un tel recours était conforme à la Constitution à la condition qu'il soit subordonné au consentement de l'étranger. Or c'est exactement ce que le texte supprime. Toutes ces dispositions anticonstitutionnelles illustrent la dangerosité d'un tel texte pour notre démocratie, d'autant plus qu'elles sont contraires aux normes supranationales, qu'il s'agisse de la convention de Genève ou de la convention internationale des droits de l'enfant. En effet, sur ce dernier point, conformément aux obligations de la France relatives à l'intérêt supérieur des mineurs rappelées à plusieurs reprises par le Comité des droits de l'enfant des Nations unies, la Cour européenne des droits de l'homme, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Comité consultatif national d'éthique et l'Académie nationale de médecine, ce projet de loi aurait dû supprimer toute possibilité de maintenir des mineurs en zone d'attente ou en centre de rétention administrative quelle que soit leur nationalité, afin qu'ils soient admis dignement sur notre territoire et mis sous la protection de l'aide sociale à l'enfance. Je l'affirme avec force : un mineur, même étranger, n'est pas un migrant. C'est un enfant, et ce jusqu'à l'âge de sa majorité. Nous lui devons donc aide et protection, et le Sénat s'honorerait en supprimant l'article 15 relatif à la durée de placement en rétention pour cinq jours des familles, car qui dit famille dit enfants. Les mesures d'enfermement pour les majeurs posent également question, comme la facilitation de la rétention administrative, notamment des « dublinés » qui n'ont commis aucun délit, alors même que la France a déjà été condamnée à six reprises par la Cour européenne des droits de l'homme à cause de ses conditions de rétention. Autre atteinte excessive aux droits fondamentaux des demandeurs d'asile, le droit inconditionnel à l'accueil et au maintien en hébergement d'urgence de toutes les personnes au regard du seul critère de la détresse, auquel contrevient l'article 9 du présent projet de loi qui légalise la circulaire Collomb de décembre 2017 tant décriée. Hélas, la liste des principes fondamentaux remis en cause par ce projet de loi est encore longue- nous y reviendrons au cours du débat.

Nous participerons au débat, en insistant notamment sur le caractère universel du principe constitutionnel d'égalité qui ne saurait tolérer la moindre distinction entre ressortissants nationaux et ressortissants étrangers s'agissant de la garantie des droits fondamentaux attachés à la personne.

Vous l'aurez compris, nous ne partageons pas votre analyse, et je vais m'en expliquer. C'est étonnant ! La commission des lois du Sénat, après un examen minutieux du texte, propose un projet de loi amélioré, détaillé et argumenté qui, en tout état de cause, respecte le droit d'asile auquel nous sommes foncièrement attachés. En effet, le rapporteur a trouvé un juste équilibre entre l'amélioration du traitement des demandes d'asile et les conditions réalistes du droit de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, dont l'activité ne cesse de croître ces dernières années.

La réduction à quinze jours semble d'autant plus inenvisageable que l'organisation actuelle de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas optimale et mérite d'évoluer. Je souhaite également attirer votre attention sur un point particulier des apports de la commission qui me tient à coeur, celui des mineurs isolés. Je tiens à féliciter la commission pour sa prise de position sur ce sujet. L'interdiction de placement en rétention des mineurs isolés est une avancée majeure, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté l'avait d'ailleurs appelée de ses voeux. L'encadrement du placement en rétention des mineurs accompagnant leurs familles, réduit à cinq jours alors que, aujourd'hui, ces familles peuvent être placées en rétention jusqu'à trente jours, est également une avancée majeure en termes d'humanité. Ces décisions courageuses étaient nécessaires pour protéger les plus vulnérables, et je tiens à en féliciter notre rapporteur. Pour ces différents motifs, mon groupe ne considère pas que ce texte soulève des difficultés constitutionnelles, et votera donc contre la présente motion Plus largement, je veux revenir sur les nombreux débats qui ont eu lieu autour de ce texte, et plus généralement, concernant la réforme de notre politique migratoire. Les termes « dignité » et « respect des droits fondamentaux » sont souvent évoqués. Pourtant, n'est-ce pas dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes que nous souhaitons mieux maîtriser les flux migratoires, afin de mieux intégrer ces femmes et ces hommes qui fuient leur pays ? N'est-ce pas dans cette même optique que nous avons soutenu l'État lors du démantèlement de la lande de Calais qui a permis, je le rappelle, de mettre à l'abri des milliers de personnes dans des centres d'hébergement offrant des conditions d'accueil dignes ? N'est-ce pas dans cette même optique encore que la petite commune de Merlimont-dont j'ai été maire-, située à quatre-vingts kilomètres de Calais, a accueilli à deux reprises, comme d'autres collectivités du territoire, des mineurs qui ont été extraits des camps de fortune où les conditions de vie étaient inacceptables ? Je me suis rendu plusieurs fois sur le terrain, tout comme certains collègues ici présents- je salue d'ailleurs le travail de François-Noël Buffet, avec qui je suis allé à Calais et à Grande-Synthe. Ces visites nous ont permis de mieux appréhender la problématique migratoire sur le territoire : la situation humanitaire, la présence et le mode de fonctionnement des associations, les actions des activistes, tout comme l'organisation des passeurs. Lors de ces déplacements, j'ai pu échanger avec les élus des communes concernées, souvent désemparés devant l'ampleur de la crise, avec les riverains, partagés entre incompréhension, sollicitude et résignation parfois, avec les services de l'État présents pour conseiller les migrants, avec les associations qui leur viennent en aide, avec les forces de l'ordre qui font un travail remarquable sur le terrain. À chaque fois, j'en suis ressorti différent, bien évidemment marqué par la situation humanitaire et la détresse dans laquelle se trouvent ces personnes qui ont quitté leur pays, pour certaines leur famille, leurs attaches, la plupart pour rejoindre l'Angleterre à tout prix, parfois même au péril de leur vie. Comment, madame Assassi, ne pas être bouleversé quand vous voyez ces femmes, ces hommes, pis, ces enfants attendre un passage inespéré vers l'Angleterre, ce pays dont on leur a tant vanté les mérites ? En ce sens, la loi en vigueur sur laquelle nous, parlementaires, ne cessons de travailler pour la faire évoluer ne répond pas à la réalité actuelle du terrain. Le projet de loi présenté par le Gouvernement et le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale n'y répondent pas complètement non plus. Notre pays doit avoir le courage de fixer clairement une politique migratoire crédible et cohérente, afin de mieux accueillir et de mieux intégrer les demandeurs d'asile, le tout, monsieur le rapporteur, madame la ministre, dans un cadre européen clarifié, apaisé et solidaire. Je rejoins donc mes collègues de la commission des lois qui ont effectué un travail important en proposant un contre-projet fourni et argumenté. de loi proposé par le Gouvernement et voté par l'Assemblée nationale ne permet pas toutes les avancées dont notre pays a tant besoin, alors qu'un tel texte doit permettre à la France d'assumer une politique migratoire ambitieuse. À ce titre, la commission des lois a adopté plusieurs mesures primordiales que je ne citerai pas en totalité- mes collègues les ont déjà développées pour la plupart, ou les développeront au cours du débat. Je pense, Je pense, bien évidemment, à l'organisation au Parlement d'un débat annuel sur la gestion des flux migratoires, à la transformation de l'aide médicale de l'État en aide médicale d'urgence centrée sur les maladies graves, la grossesse, ainsi bien sûr que la médecine préventive. Je pense aussi aux collectivités territoriales. Les élus locaux directement concernés me disent souvent se sentir démunis face à cette crise migratoire. Leur voix n'est malheureusement que trop peu entendue, alors que leur place dans les réflexions à mener est tout à fait légitime. Les sanctions à l'encontre de ceux qui enfreignent nos règles doivent être renforcées, et les mesures d'éloignement envers les déboutés doivent être plus efficaces. En ce sens, toute décision définitive de rejet d'une demande d'asile doit valoir obligation de quitter le territoire français. Je salue également la décision de réduire le nombre de visas accordés aux pays les moins coopératifs pour délivrer les laissez-passer consulaires indispensables à l'éloignement des personnes en situation irrégulière. En tant que sénateur du Pas-de-Calais, je souhaite également revenir sur la situation particulière de mon département, point de chute de centaines, voire de milliers- il en fut -de personnes fuyant leur pays. Depuis le démantèlement de la lande, la situation calaisienne a certes évolué. La preuve en est qu'il y a quelques jours a été inauguré le site naturel des Deux Mers en lieu et place de l'ancienne lande. Cette renaturation montre qu'une page s'est tournée sur ce site, qui a malheureusement attiré les yeux du monde entier. Toutefois, ne nous leurrons pas, la problématique migratoire n'a pas totalement disparu pour autant : en témoignent la mobilisation des forces de l'ordre sur le terrain et les incidents récurrents. J'ai, par exemple, été interpellé par les transporteurs routiers de marchandises qui effectuent du transport transmanche. Ces professionnels subissent toujours les conséquences de la présence migratoire à Calais. Les intrusions sur les sites des entreprises et la dégradation des matériels ou des marchandises transportées n'ont absolument pas cessé. Cette situation crée un réel sentiment d'insécurité chez les chauffeurs routiers. De plus, elle entraîne des coûts financiers importants pour les entreprises qui voient leur matériel ou leurs marchandises dégradés, sans compter les amendes infligées en cas de découverte d'un ou plusieurs migrants dans un camion contrôlé en France par les forces de l'ordre britanniques. Enfin, les conséquences financières et économiques sur ce territoire continuent à se faire ressentir. L'État affirme oeuvrer afin qu'aucun point de fixation ne se crée. Toutefois, je m'interroge, madame la ministre, sur la vision à long terme du Gouvernement pour le Calaisis. Comme je l'ai affirmé il y a plus d'un an, si nous ne pouvons fermer la porte aux personnes demandant légitimement l'asile, il me semble primordial de redéfinir notre politique migratoire dans un cadre européen propice

de la commission : le maintien du délai de recours devant la CNDA à trente jours, la protection des mineurs en rétention, ainsi que la nécessité dans les politiques de fermeté et d'éloignement de garantir à l'ensemble des

Chacune des mesures que vous évoquez a été soigneusement pesée pour s'assurer de sa pleine conformité avec l'ensemble des droits de la défense constitutionnellement et conventionnellement garantis. Vous n'allez pas de constater que chacune des mesures dont vous contestez la conformité aux normes supérieures existe de façon équivalente chez bon nombre de nos voisins européens. Vous critiquez par exemple, madame la sénatrice, une disposition qui instaurerait une justice expéditive. Or il ne faut pas confondre le délai pour saisir la justice, qui est de quinze jours dans une dizaine de pays européens, et le délai pour juger, qui est le seul sur la base duquel on pourrait critiquer une justice expéditive. Quant à la prise en compte des vulnérabilités particulières des demandeurs d'asile, et plus largement des étrangers, je ne peux que rappeler la mobilisation du Gouvernement à ce sujet. Ainsi, nous menons une action qui vise à la fois à concentrer nos efforts sur les publics les plus vulnérables et à prendre en compte la vulnérabilité des personnes à toutes les étapes de la procédure. Pour ce qui concerne les publics les plus vulnérables, nous portons une attention particulière aux femmes, notamment aux femmes victimes de violences. Comme vous le savez, le texte contient plusieurs dispositions sur ce sujet, mais au-delà, nous allons développer des structures d'hébergement spécialisées pour leur prise en charge, particulièrement pour leur soutien psychologique. En 2018, sept structures seront ainsi créées. Par ailleurs, ces dispositifs seront également étendus aux membres de la communauté LGBT. Notre action envers les personnes les plus vulnérables s'étend aussi au-delà de notre territoire à travers la réinstallation des réfugiés en fort besoin de protection. Vous savez que l'objectif est d'en accueillir 10 000 d'ici à 2019. Il s'agit, par exemple, de réfugiés soudanais du Darfour victimes de persécutions, mais aussi de personnes, notamment des femmes, victimes je suis particulièrement attachée à ce que la vulnérabilité des personnes soit prise en compte à toutes les étapes de la procédure d'asile. dès le premier accueil au moment de l'enregistrement de la demande d'asile, le repérage de la vulnérabilité est au coeur du dispositif des CAES que nous déployons sur le territoire. Ces informations sont précieuses pour l'enregistrement des demandes auprès Par ailleurs, l'orientation directive des demandeurs dans le dispositif national d'asile prendra en compte la vulnérabilité des personnes. Comme je l'indiquais précédemment, les publics les plus vulnérables seront en priorité orientés vers les structures assurant une prise en charge spécifique de leur vulnérabilité. En outre, nous allons prochainement lancer un appel à projets visant à développer la prise en charge psychologique et sanitaire des migrants. Enfin, la vulnérabilité fait l'objet d'une prise en compte spécifique lors de l'instruction des demandes par l'OFPRA et la CNDA. Ainsi les personnels qui instruisent ces dossiers disposent de formations spécifiques pour déceler la vulnérabilité psychologique, et des groupes de travail thématiques ont été mis en place à l'OFPRA depuis 2013. vous le voyez, la mobilisation du Gouvernement est totale pour que la maîtrise de l'immigration se fasse dans un cadre respectueux de la dignité et des droits de chacun. La parole

apportée. La liste des principes fondamentaux remis en cause par ce projet de loi était pourtant encore longue : du droit au procès équitable bafoué au principe d'unité familiale amoindri- plus encore par la commission des lois du Sénat -, en passant par la rupture d'égalité de traitement des citoyens, avec une justice au rabais institutionnalisée outre-mer et à Mayotte en particulier, notre démocratie ne sortira pas grandie de cette prévalence de la suspicion et de la répression quant au respect et à l'effectivité des droits et des principes fondamentaux de la République. M. Macron a poursuivi un bien triste chemin depuis le sommet européen qui s'est tenu il y a un an à quelques jours près, à l'issue duquel, tenant une conférence de presse avec Mme Merkel il déclarait : « Nous devons accueillir des réfugiés, c'est notre devoir et notre honneur. Lorsque l'est passé à sept kilomètres de nos côtes, chassé d'Italie par un ministre de l'intérieur néofasciste, le chef de l'État avait semble-t-il oublié ces belles paroles. On dit souvent que le Président de la République fait ce qu'il dit, ce qu'il a promis. Si certaines dispositions avaient été annoncées, rien ne permettait de prévoir la violence de la politique menée par ce gouvernement ainsi que la violence de certains propos tenus en certaines circonstances. Un avant-goût amer de ce projet de loi avait été annoncé par vos circulaires de décembre relatives au recensement administratif dans les centres d'hébergement et à la demande faite aux préfets d'accroître les reconduites à la frontière. Avec ces textes, vous avez donné le la. L'historien Patrick Weil a déclaré à ce sujet : « Aucun gouvernement depuis la Deuxième Guerre mondiale n'avait osé aller jusque-là ». Évoquant le futur projet de loi, il poursuivait [de loi] s'inscrit dans cette lignée, ce sera une régression dramatique. » Nous sommes aujourd'hui face à cette régression dramatique contraire à nos principes fondamentaux et à la tradition républicaine de notre pays

Nous ne devons pas céder à cette facilité dangereuse, qui tend à dresser les peuples les uns contre les autres dans un débat démocratique. Que vous l'admettiez ou non, vous jouez sur la peur de l'autre, sur l'individualisme, comme d'autres l'ont fait bien mieux auparavant.

de très nombreux sénateurs le sont, preuve s'il en est que le Sénat est vraiment une institution indispensable à la vie démocratique.

a trait à la durée de rétention. Selon un scénario assez complexe, celle-ci, qui était déjà de 45 jours, alors que chacun sait qu'au-delà de douze jours elle n'a plus d'utilité, avait été doublée dans le projet de loi gouvernemental, pour des raisons que nous avons comprises lorsque le ministre Collomb a dit qu'il redoutait le des migrants, pour finalement être réduite de nouveau à 45 jours par la commission des lois, mais augmentée à six mois pour certains

l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Nous eussions pu comprendre que le choix eût été fait pour vous de représenter la France en Allemagne. Las, M. le ministre de l'intérieur n'est pas là,

Parce que, d'abord, il n'aura pas d'efficacité- vous le savez -au regard des objectifs qu'on lui assigne.

mes chers collègues, que son texte nous ait tous marqués. Elle a évoqué ces que nous avons accueillis généreusement, sans compter, parce qu'il fallait le faire, et tant d'autres tragédies de l'histoire où la loi essentielle et première est celle de l'humanité. Je songe à ce dessin de Plantu dans où l'on voit un bateau au milieu de la Méditerranée et, sur ce bateau, un fonctionnaire qui fait son travail : les affamés, leur dit-il, levez le doigt ! De manière qu'on puisse distinguer ceux qui crèvent de faim et ceux qui ont la légitimité pour être accueillis ... Je comprends ce discours, mais je perçois ce qu'il a de tragique. La réalité, c'est que la mer Méditerranée, où est née la civilisation, est devenue un cimetière à ciel ouvert.

qu'on ne pouvait accueillir toute la misère du monde, et il a eu raison ; il a dit, en plus, qu'il fallait que la France en prenne toute sa part, et il a eu raison aussi.

ces deux jours de triste silence de la France, avant de tardifs efforts diplomatiques. Fallait-il tout ce temps pour comprendre que la Corse est plus proche de la Sardaigne que de l'Espagne

est, une fois encore, de tenter de rassurer ce qu'on appelle l'opinion contre l'ancestrale peur de l'étranger. Madame la ministre, vous devriez retirer ce texte aussi parce qu'il ne consacre pas une seule phrase à la question européenne- pas même un mot, comme M. le rapporteur l'a expliqué. Il nous faut pourtant mener un combat commun, un combat de la France, contre l'Europe de la fermeture, de l'exclusion et de la xénophobie qui progresse à grands pas. promouvoir une autre philosophie européenne, une autre conception de l'Europe : une Europe qui lutte plus efficacement contre les passeurs, pour la maîtrise des frontières et pour une vraie coopération avec les pays d'origine. Renouer les liens avec l'Afrique, reconstruire l'Euroméditerranée : il y a tant à faire ! Mais votre texte, madame la

et raccourcir les délais de recours change quoi que ce soit au fait que, aujourd'hui, 13 % des OQTF donnent lieu à exécution

aussi ne pas entendre, madame la ministre, l'avis extrêmement précis du Conseil d'État, qui vous demande : pourquoi ne pas avoir évalué l'effet des lois de 2015 et 2016 avant que de faire cette nouvelle loi ? Conseil d'État ne trouve pas dans le contenu de ce texte le reflet d'une stratégie prenant en compte l'immigration et les faits migratoires tels qu'ils sont aujourd'hui et tels qu'ils se dérouleront demain.

faire, d'après vous ? Je sais, madame la ministre, que vous le savez profondément : sur cette terre, on a besoin de tout le monde. Et il arrive en effet que des sans-papiers,

j'ai tâché d'imaginer ce qu'aurait dit l'un de nos grands ancêtres, ici au Sénat et à la Chambre des pairs, Victor Hugo, s'il avait dû décrire ce qui se passe aujourd'hui en mer Méditerranée.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au nom des sénateurs du groupe Les Républicains, permettez-moi de détailler les raisons pour lesquelles nous estimons qu'il est nécessaire

grâce aux nombreuses heures de travail consacrées à son examen par la commission des lois et son rapporteur, notre collègue François-Noël Buffet, dont je salue l'investissement et la détermination, ce projet de loi, qui n'était à l'origine que le résultat d'un compromis bancal entre la jambe droite et la jambe gauche de la majorité présidentielle, est devenu un outil plus efficace, plus concret et plus solide, que nous entendons faire servir à la maîtrise de l'immigration en France, notamment à la lutte contre l'immigration irrégulière. Partons d'un constat que nul ne peut contester, pour peu qu'il fasse preuve de clairvoyance et de bonne foi : nos compatriotes n'acceptent plus de voir l'État baisser les bras face aux flux migratoires sous le poids desquels croulent nos services chargés du traitement des demandes d'asile et du contrôle de l'immigration. En deux ans, en 2015 et 2016, 2,3 millions de migrants sont entrés illégalement dans l'espace Schengen, contre 100 000 en moyenne les années précédentes. Cette pression migratoire est toujours extrêmement soutenue en France, et les flux à l'échelon européen se réorganisent sans se tarir, en raison de la montée des conflits armés, de la pauvreté persistante dans les pays en développement et des conséquences environnementales du réchauffement climatique. Sommes-nous prêts, mes chers collègues, à affronter un tel défi ? De toute évidence, non. Il est donc de notre devoir de nous y préparer en renforçant nos exigences et nos critères d'admission en France, afin que nos enfants et petits-enfants puissent vivre dans un pays disposant toujours de la maîtrise de son propre destin. En 2017, la France a admis 260 000 nouveaux immigrés réguliers, le record des quarante dernières années. En parallèle, dans le cadre de la loi de finances pour 2018, le budget de la lutte contre l'immigration irrégulière a diminué de 7 %. Les fonds consacrés à l'aide médicale de l'État, eux, ont augmenté dans le même temps de 13

comme sur de nombreux sujets, la montagne gouvernementale a accouché d'une souris. En effet, face aux enjeux majeurs que je viens d'évoquer, le texte proposé par le Gouvernement et adopté par sa majorité à l'Assemblée nationale est une bien faible réponse. Sacrifiant toute fermeté et tout pragmatisme à la nécessité de ne pas heurter son aile gauche, le Gouvernement présente un texte technique qui n'apporte en réalité aucune solution crédible aux problèmes d'aujourd'hui, encore moins à ceux de demain. Demain, c'est l'horizon qu'il nous faut regarder, si nous voulons mener une réforme véritablement efficace pour les générations futures. Hélas, le Gouvernement n'a pas souhaité traiter ces problèmes en profondeur. Ce texte, focalisé sur le droit d'asile, dont la nécessité ne fait absolument aucun débat, ne changera rien au véritable problème de fond : la faiblesse des moyens financiers et humains alloués à la lutte contre l'immigration irrégulière. En 2015, seuls quatre immigrés en situation irrégulière sur cent ont été effectivement reconduits à la frontière. Pendant ce temps, des milliers de demandeurs d'asile sont accueillis par l'État, parfois dans des gymnases, dans l'attente de l'examen de leur situation administrative. Enfin, le texte gouvernemental s'avère extrêmement permissif en ce qui concerne la réunification familiale à l'égard des frères et soeurs des réfugiés mineurs. Une disposition que nous avons bien sûr supprimée au sein de la commission des lois, tant elle sème les germes de drames à venir sur le plan humanitaire combien de mineurs seront-ils envoyés seuls, au mépris des risques, dans les mains des passeurs, sur les routes et par-delà les mers, dans l'espoir d'atteindre la France, d'où ils pourront faire venir leurs frères et soeurs ? Prenons conscience tous ensemble, pour l'accepter, de la réalité des lourdes charges financières qui incombent aux départements en matière de prise en charge des mineurs non accompagnés. Pour citer un exemple que je connais bien, en 2010, le département du Val-d'Oise prenait en charge 80 80 mineurs isolés, pour un coût de 3 millions d'euros ; en 2018, il en accueille 640, pour un montant de 43 millions d'euros. La commission des lois s'est donc pleinement saisie de ce texte et l'a profondément modifié, à la suite des très nombreuses auditions des responsables associatifs et des représentants des services de l'État que nous avons menées. Ainsi, nous proposons au Sénat de refuser le statut de réfugié à ceux qui constitueraient une menace grave pour la sûreté de l'État ; de refuser l'extension de la réunification familiale aux frères et soeurs des réfugiés mineurs ; de créer un fichier national des mineurs ; de donner à toute décision définitive de rejet d'une demande d'asile valeur d'obligation de quitter le territoire. Non, ces dispositions ne suffiront pas à régler définitivement la question de l'immigration en France. Mais, oui, face au manque de volonté du Gouvernement, elles permettront de pallier un certain nombre de défaillances de notre système d'asile et d'immigration et d'affirmer la détermination du Sénat à agir. Ce projet de loi, largement amendé par notre assemblée, constituera notre appel en faveur d'une véritable politique migratoire en France. C'est pourquoi le groupe Les Républicains vous appelle, mes chers collègues, à ne

du Gouvernement ? Le groupe socialiste et républicain conteste la nécessité du projet de loi, qui serait une énième modification du droit des étrangers, opérée sans qu'on ait pu évaluer l'efficacité des modifications législatives antérieures.

Ce sont ces constats qui justifient le projet de loi qui vous est soumis. Les grands objectifs du Gouvernement sont de traiter les demandes d'asile en six mois et de tirer toutes les conséquences en matière d'éloignement pour renforcer effectivement l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière, mais aussi de mieux intégrer les personnes qui ont vocation à rester sur le territoire- je crois que nous sommes tous d'accord avec cela. Ces objectifs sont, contrairement à ce que vous affirmez, à la hauteur des défis auxquels nous faisons face ils visent à permettre une réelle maîtrise de l'immigration, dans le respect des droits des personnes. Face au constat du durcissement des politiques migratoires à l'échelle européenne- vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe dans un certain nombre de pays,

ont pourtant longuement occupés dans cet hémicycle. Je dois d'ailleurs dire que mon groupe a alors vécu de grands moments de solitude ... Mais sachez que l'expérience quotidienne des professionnels et des bénévoles au contact des demandeurs d'asile et des étrangers nous livre déjà un état des lieux loin d'être réjouissant. Et pour cause : en matière de délais d'examen des demandes d'asile,

Le scrutin est ouvert.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, à peine trois ans ont passé depuis la dernière réforme de l'asile et la dernière refonte du droit des étrangers, toutes deux menées par l'ancienne majorité trois années qui n'auront permis ni de faire un bilan précis de l'efficacité des mesures votées ni d'élaborer une véritable politique migratoire, ambitieuse et rationnelle. Le texte que nous examinons en procédure accélérée est au moins le vingt-neuvième depuis la fin des années Notre législation tourne à vide. Elle ne semble avoir qu'une boussole : le Rassemblement national. Or ce n'est pas en s'alignant sur les thèmes du RN, ex-FN, que l'on réussira à faire reculer les votes en sa faveur, Jacques Toubon lui-même. On nous promettait un nouveau monde. Le candidat Macron rappelait, en janvier 2017 à Berlin : « On ne peut pas revoir nos valeurs à l'aune des risques du monde

Pour nos dirigeants, les exilés ne sont que des encombrants, un flux à gérer, un chiffre à réduire. Chacun sait que la prise en charge équitable des exilés par les pays de l'Union européenne est la seule issue. Mais ce n'est pas parce qu'il est urgent de mettre en oeuvre une vraie politique européenne que la France doit tout s'autoriser. Lisez le rapport 2018 de la Contrôleur général des lieux de privation de liberté, sur ce qui se passe à Menton : « La prise en charge quotidienne de personnes étrangères s'effectue dans des conditions indignes et irrespectueuses de leurs droits. » Lisez le rapport d'Oxfam de ce mois sur la situation des exilés à la frontière franco-italienne. Il est aussi accablant pour la France que pour l'Italie. Heureusement, notre pays a ses délinquants solidaires, ses associatifs, ses citoyens de bonne volonté qui, contre une opinion publique remontée, portent secours à ces sans-rien que d'aucuns rêveraient de voir tout simplement disparaître sous leur talon. Une majorité de nos compatriotes était contre l'accueil de l'dans l'un de nos ports. Et alors ? Faut-il les en féliciter ? féliciter le peuple espagnol d'avoir épaulé son gouvernement, plus de 1 000 bénévoles s'étant dévoués pour accueillir les rescapés Quel contraste avec notre commission des lois, qui a même trouvé le moyen de supprimer le petit assouplissement que l'Assemblée nationale avait apporté en faveur des aidants au transport, en limitant à la marge notre définition du délit de solidarité Décidément, rien ne doit brider l'oeuvre de maltraitance de ce gouvernement. À l'intention de sa droite, de la droite dure et même de l'extrême droite, l'exécutif fait miroiter un durcissement législatif susceptible de favoriser une augmentation des expulsions de migrants économiques la nuance, cher collègue ! Or les législateurs que nous sommes ne peuvent ignorer que le budget voté il y a quelques mois ne prévoit pas de moyens supplémentaires

dans le langage courant, que des « migrants ». Ce glissement lexical contribue à semer la confusion entre immigration économique et accueil des réfugiés. Il revient à faire oublier les conventions internationales que nous avons signées. Les « migrants », ceux de l'et de tous les bateaux affrontant une Méditerranée meurtrière ; les « migrants dont on retrouve le corps sans vie dans les Alpes après la fonte des neiges ; ces mêmes « migrants » de Calais et de la porte de la Chapelle sont des hommes, des femmes et des enfants, nos semblables

définition européenne du droit d'asile ; le dispositif de reconnaissance mutuelle des jugements statuant sur les demandes d'asile qui pouvait être espéré entre les États ; l'aide au développement qui été

en Europe de l'Est. Enfin- vous le savez également -, l'Europe est attaquée dans sa souveraineté, dans sa capacité d'action politique et économique, par des pays adeptes des rapports de force, voir par des États historiquement amis. C'est dire que nous ne pouvons pas nous permettre un désaccord de plus, sur le sujet migratoire. C'est dire aussi que le

Notre pays n'assume pas sa responsabilité ou ne fait pas en sorte que les choses se passent si efficacement que l'on pourrait le souhaiter, pour les personnes que nous avons accepté d'accueillir sur le territoire et qui bénéficient

par le juge des libertés et de la détention. Nous prenons en compte le besoin, exprimé par le Gouvernement, de pouvoir négocier avec les États des laissez-passer consulaires et de disposer de

en interdisant l'enfermement des enfants. Enfin, nous défendrons un droit à l'autonomie des demandeurs d'asile en affirmant un droit à la formation linguistique et au travail, dès que les directives européennes le permettront.

parce que nous ne sommes pas résilients, affaiblir tous nos voisins, les faire évoluer vers des systèmes qui ne sont pas conformes à nos valeurs ? Ce débat est essentiel. Il est essentiel pour l'avenir de l'Europe.

Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la crise des migrants est un drame européen. texte, à lui seul, ne permettra pas de résoudre une question qui est véritablement existentielle pour l'Union européenne. On pourra l'utiliser à des fins politiques, l'accuser d'être laxiste, ou encore d'être trop dur. Mais il faut garder à l'esprit que l'essentiel se joue ailleurs ; l'essentiel se joue à Bruxelles. Hélas, la politique commune de l'asile et de l'immigration a jusque-là été un échec patent. Construite pour des flux faibles, elle n'a pas résisté à un afflux massif de réfugiés politiques et économiques. Le système Dublin III, adopté dans l'urgence, s'est révélé impuissant à enrayer le phénomène. l'Union européenne est aujourd'hui placée face à un dilemme existentiel : se réformer efficacement ou voir la solidarité des États membres se déliter jour après jour. Le Conseil européen des 28 et 29 juin devra prendre des positions claires. effectivement, est aussi une crise de solidarité des États membres. Les populistes de tous bords surfent sur la vague migratoire pour remettre en question le projet européen. L'exemple dramatique de l'illustre ce cynisme destructeur, qui met en péril la cohésion des Européens. J'ajoute, mes chers collègues, que l'échelle européenne est également la plus pertinente pour définir une politique commune d'attraction des talents, à la mesure de celle qui se pratique, par exemple aux États-Unis, avec la, ou au Canada. L'extension du passeport talent, prévue dans le projet de loi, est une bonne chose. Nous devons nous donner les moyens d'attirer les scientifiques, les artistes, les chefs d'entreprise les plus talentueux du monde pour faire rayonner notre pays et notre continent. L'Union européenne ne deviendra pas « l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde », pour reprendre les termes de la stratégie de Lisbonne, sans s'ouvrir aux compétences du monde entier. Madame la ministre, mes chers collègues, que ceux qui réclament moins d'Europe et, en même temps, le règlement de la crise des migrants regardent la vérité en face : la solution au problème des migrations et de l'asile sera politique, elle sera européenne, elle sera collaborative ou elle ne sera pas

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'actualité fait une fois de plus écho à nos débats.

Bien qu'il ne concerne qu'une partie très minoritaire de la population en France, le droit des étrangers a été très régulièrement modifié depuis les années quatre-vingt, avec pas moins de vingt-neuf textes sur le sujet. Comment expliquer cette surreprésentation législative ? La première raison que l'on peut avancer est l'inadaptation de la méthode retenue. L'arrivée d'étrangers sur le territoire national continue d'être abordée comme un phénomène conjoncturel, une crise passagère, alors que, compte tenu de l'évolution structurelle des flux migratoires et de la permanence des conflits suscitant l'exil- Irak, Syrie, Afghanistan, pour ne citer que ces pays -, il est indispensable d'adopter une démarche plus prospective. Il faut totalement repenser notre système d'accueil et d'intégration, de l'hébergement d'urgence à l'exécution des décisions administratives. Partout en Europe, le populisme gagne du terrain en se nourrissant de la question migratoire. Une approche globale est donc absolument nécessaire, si l'on veut que les Français ne perçoivent pas notre politique d'accueil et d'intégration comme une charge déraisonnable et contraire à leurs intérêts.

À ce titre, nous sommes nombreux à penser que ce débat se serait déroulé dans un contexte plus satisfaisant s'il s'était inscrit dans la continuité de mesures destinées à restaurer la justice sociale dans l'ensemble des territoires de la République. En effet, chaque réforme du droit des étrangers et des demandeurs d'asile est essentiellement politique et ne peut être présentée comme une simple réponse à une crise ou une mise en conformité avec le droit européen ou international. Malgré les textes à valeur supralégislative, l'accueil de réfugiés, la reconnaissance d'un droit au séjour ou l'attribution de la nationalité française restent des décisions unilatérales. Chaque modification de ces droits est un miroir tendu vers notre société, une invitation à redéfinir collectivement ce que nous sommes. Dans cet effort de définition, notre histoire devrait nous guider autant que les défis contemporains qui surgissent. Dans un passé pas si lointain, réfugiés et immigrés étaient perçus comme des vecteurs de rayonnement de la France dans le monde. Cela me conduit à la seconde cause de la multiplication des lois relatives aux droits des étrangers : l'interdépendance de nos sociétés contemporaines. Lorsque l'on se place dans une logique de régulation des flux migratoires, et non plus seulement d'accueil ou d'intégration, la coopération avec l'ensemble des États devient une nécessité absolue. Malgré notre impuissance à imposer à nos partenaires la généralisation de pièces d'identité, ce qui faciliterait considérablement la gestion de la politique migratoire, il faut se garder de vouloir apporter des solutions législatives affectant les libertés fondamentales sans s'assurer au préalable de leur efficacité. Je pense tout particulièrement au problème des laissez-passer consulaires. L'étude d'impact produite par le Gouvernement est muette sur ce point-là. La solution législative proposée par le rapporteur, consistant à conditionner la délivrance de visas individuels à la propension des États à délivrer des laissez-passer, bien qu'intéressante, nous paraît trop contraignante pour nos services diplomatiques. L'interdépendance de nos sociétés nous impose également de dresser un état des lieux approfondi de notre politique de codéveloppement et de nous départir d'idées préconçues. Les trajectoires de certains États, comme le Kenya, où l'immigration a été considérablement réduite, doivent être examinées de plus près, afin d'inspirer des solutions durables. Madame la ministre, mes chers collègues, après ces constats, vous l'aurez compris, le texte amendé et singulièrement durci par la commission des lois n'obtiendra pas l'adhésion du Même en reconnaissant les différentes pressions migratoires existant d'un territoire à un autre, le projet de loi n'y apporte pas de réponse. En particulier, la situation des outre-mer est largement sous-estimée. Je pense notamment à Mayotte et à la Guyane, mais également à mon territoire, Saint-Martin, qui doivent faire face à un afflux important de migrants au regard de leur taille ou de leur population, fragilisant fortement les équilibres locaux. Un seul article est consacré au schéma national d'orientation et ne permettra pas de pallier les difficultés chroniques dans les services publics régaliens ou de garantir des solutions d'hébergement d'urgence effectives. De même, l'absence de dispositions contraignantes relatives à la question des futurs réfugiés climatiques, tout comme le nombre limité des mesures relatives à l'intégration sont symptomatiques de la faiblesse de la démarche prospective que j'évoquais précédemment. Ce texte ne présente pas davantage de solutions pour lutter contre la traite d'êtres humains à laquelle se livrent les passeurs. Nous proposerons donc une série d'amendements, visant plusieurs objectifs. L'amélioration de la protection des mineurs, même accompagnés. Une réflexion pourrait s'ouvrir sur les moyens d'offrir un accueil plus adapté aux mineurs isolés étrangers et sur les possibilités de recourir, pour eux, à l'adoption. La facilitation du codéveloppement. Le but serait de faire émerger des alternatives politiques partout où les États vacillent. D'autres amendements, inspirés de nos visites et de nos auditions, tendront à garantir une plus grande qualité d'interprétariat et à mieux répartir les différents publics en centre de rétention administrative. Enfin, nous proposerons de confier un rôle plus important aux élus locaux dans la procédure de régularisation administrative, eux qui sont souvent les premiers témoins de la volonté d'intégration de chacun. À titre d'illustration, je suggère la création d'un office des migrations à Saint-Martin, pour mieux coordonner la délivrance des titres de séjour et de travail. je reste convaincu que notre pays, sixième puissance économique mondiale, dispose des ressources intellectuelles et matérielles pour mieux répondre aux défis posés par ce siècle, pour entraîner avec lui ses partenaires européens et influer sur le reste du monde. Dans sa forme actuelle, le groupe du RDSE s'opposera unanimement à l'adoption de ce projet de loi.

nous soutiendrons celle qui est portée dans ce texte, avec un double objectif : rester fermement engagés pour l'accueil des réfugiés politiques et renforcer notre capacité à maîtriser l'immigration économique.

Cette distinction est pourtant nécessaire et équitable. Faute de la formuler avec clarté, on facilite l'excès contraire, le choix des populistes xénophobes qui, eux, veulent refuser tous les réfugiés et tous les immigrés. C'est l'opinion exprimée aujourd'hui, souvent avec brutalité, par plusieurs gouvernements de l'Union européenne.

Ayons pourtant claire à l'esprit une réalité déplaisante. Les traités fondant la construction européenne, telle qu'elle est, traités conclus entre vingt-huit démocraties, ne donnent pas compétence à l'Union européenne pour statuer sur le droit pour les étrangers d'entrer sur le sol européen. C'est une matière de souveraineté nationale et nous ne pourrons progresser vers une action harmonisée que par de nouveaux accords, qui exigeront le consentement de vingt-sept gouvernements et de vingt-sept parlements exprimant aujourd'hui des approches très différentes. L'agence européenne de l'asile et du séjour proposée par le président Emmanuel Macron exigera un effort, que nous devons soutenir sans nous bercer d'illusions. Pour conclure des accords nouveaux, on en passera nécessairement par des compromis difficiles et sans doute partiels, unissant une partie, seulement, de l'Union européenne. Cela ne peut par conséquent pas nous dispenser, aujourd'hui, de débattre et de décider pour notre propre droit. Donc oui, il faut adopter les nouvelles dispositions proposées, qui statuent sur la situation réelle ! Il faut prévoir des outils améliorés, pour accélérer l'attribution du titre de réfugié à toute personne apportant la justification des persécutions qu'elle encourt du fait d'une crise ou d'un conflit dans sa région d'origine. Cette reconnaissance, et le projet de loi le permet, doit se faire en donnant à chacun toutes les garanties du droit pour plaider sa cause dans un processus équitable.

Laisser cette question irrésolue, ce qui me semble être la tentation d'une partie des adversaires du texte, équivaut- j'y insiste -à dénaturer le droit d'asile, qui appartient à notre tradition protectrice issue des Lumières et de la Révolution française.

Accepter une ouverture non maîtrisée à une immigration économique, dans notre contexte démographique et social, c'est en réalité se résigner à des situations de marginalité sociale et d'économie grise, qui porteraient- et portent déjà -gravement atteinte à notre cohésion sociale. Je ne parle même pas du rôle des filières mafieuses et meurtrières qui s'enrichissent dans ces trafics

l'amendement de notre collègue Thani Mohamed Soilihi relatif au droit de la nationalité spécifique à Mayotte. Notre débat sera par conséquent un test de volonté politique face au réel, avons à approfondir les modalités au cours du débat des articles. Adopter un texte d'équilibre et de clarification de nos règles, en soutenant une politique européenne et internationale de rééquilibrage et de maîtrise des mouvements migratoires, c'est une prise de responsabilité. Mon groupe l'assume avec détermination

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, qui représentons-nous ? Qui sommes-nous ?

Ne vous faites pas d'illusions ! Les fractures sociales seront d'autant plus nettes que nous ne serons pas maîtres de la situation et capables de nous imposer. Et je ne veux pas que la France soit l'Autriche ! La parole est

Au vu des difficultés majeures que notre pays rencontre en raison des flux migratoires, nous aurions aimé trouver, dans le projet de loi initial pour une immigration la traduction d'une stratégie, d'une vision, d'une politique s'appuyant sur le constat, lucide et éclairé, des défis à relever. Car ce ne sont pas de simples mesures d'ajustement, de petits aménagements procéduraux ou encore de dispositions purement techniques dont la France a besoin La commission des lois du Sénat l'a bien compris, puisqu'elle a proposé un contre-projet réaliste, reposant sur un équilibre entre fermeté et humanité. Je tiens donc à saluer le travail de réécriture qui a été effectué. Parmi les nombreuses dispositions adoptées, apportant des réponses cohérentes à des difficultés majeures, je veux en souligner quelques-unes, comme le remplacement de l'aide médicale de l'État par une aide médicale d'urgence, le renforcement des conditions du regroupement familial ou la réintroduction de la visite médicale des étudiants étrangers, afin de répondre à un grave enjeu de santé publique. La commission des lois a également interdit le placement en rétention des mineurs isolés et encadré rigoureusement celui des mineurs accompagnant leur famille. Elle a supprimé la circulaire Valls, précisant les conditions d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière, qui avait permis, sur la période 2012 à 2017, la régularisation de plus de 180 000 ressortissants étrangers séjournant illégalement en France. Or, si l'acquisition de la nationalité française vient couronner un processus d'intégration

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'immigration est un sujet dont nous parlons beaucoup, mais sur lequel nous faisons encore assez peu. Pourtant, l'actualité est là, sous nos yeux des frontières allégrement franchies, des navires traversant la Méditerranée, des pays débordés et des opinions publiques inquiètes, à qui l'on répond parfois avec condescendance ou mépris ! Ne soyons pas idylliques à propos de ces flux migratoires. Je sais qu'il existe des situations de détresse, qui peuvent émouvoir, mais il y a aussi des passeurs et des réseaux qui exploitent ces trafics sans la moindre vergogne. Il n'y a pas que des gens qui veulent tenter leur chance ; il y a aussi des mafias et des trafiquants de drogue. L'immigration sauvage intéresse aussi les profiteurs, voire les terroristes. Un pays qui maîtrise ses flux migratoires accueillera mieux ceux qui veulent s'intégrer. La France n'est pas une terre à prendre, mais un pays à aimer N'ayons pas honte d'être fermes et exigeants ! Notre pays a toujours accueilli les bonnes volontés, dont certaines ont même accepté de mourir pour lui. Ce sont curieusement ceux dont on entend le moins parler, parce qu'ils ont l'humilité de ne pas prendre nos bonnes consciences en otage. otage. Il y a aussi la cohorte de ceux qui abusent, parce que la France apparaît comme un pays qui offre une protection sociale et des allocations. Mon pays n'est pas un numéro de sécurité sociale ou un distributeur de prestations qu'il suffirait d'obtenir en cochant la case d'un formulaire Parce que le « en même temps » donne des solutions boiteuses et floues, pour ne pas dire communautaristes, en matière d'immigration, le projet de loi soumis au Sénat était inquiétant. À cet égard, je voudrais saluer le travail du président de la commission des lois, Philippe Bas, et du rapporteur François-Noël Buffet, qui n'ont pas hésité à apporter les corrections nécessaires à un texte dans lequel figuraient parfois des dispositifs irresponsables. Notre philosophie est celle de la responsabilité, non celle de l'angélisme. L'instauration d'un débat sur la politique migratoire, tout comme l'identification de nos besoins, est une mesure de bon sens. Les conditions du regroupement familial ont été restreintes l'augmentation de la durée de séjour, portée à vingt-quatre mois au lieu des douze les réfugiés, la réunification familiale ne saurait être étendue aux frères et aux soeurs. Ce problème des mineurs pénalise les départements, même Paris. les collectivités locales doivent être associées au traitement des questions relatives à l'asile : je me réjouis que la commission des lois ait prévu de les consulter pour l'élaboration des schémas régionaux d'accueil des demandeurs d'asile.

la commission des lois a demandé que toute décision définitive de rejet d'une demande d'asile soit considérée comme une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF OQTF ! Sur les questions d'immigration, nous devons être francs dans le choix des mots et éviter les contorsions qui démontrent que, même dans les esprits, on se censure ! On parle de migrants au lieu de parler de clandestins. Il est symptomatique d'employer l'expression de « délit de solidarité », alors qu'il n'y a rien d'autre qu'une violation de la loi, le soutien à une installation illégale sur le sol français. C'est de la délinquance, et rien d'autre ! Les termes existent, utilisons-les le délit d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier tel quel, et non utiliser une métaphore. Il est surprenant de voir que ceux qui s'insurgent contre l'existence de cette infraction pénale veulent à tout prix pénaliser ceux qui appellent au respect de nos frontières. Aider les clandestins, ce serait bien, mais alerter sur la porosité de nos frontières, ce serait mal ! C'est le comble de la confusion dans un pays où le terrorisme intellectuel a beaucoup sévi dans les esprits Notre tâche est lourde : il faut rassurer les Français qui sont inquiets sur ce sujet. Ceux-ci attendent de nous un message et craignent qu'il ne soit trop tard. Ils réclament des mesures fortes. Et tant mieux si c'est le Sénat qui peut leur donner cet espoir : il est le gardien de la République, mais aussi de la France et de son identité. La défense de l'une ne va pas sans l'autre ! Parce qu'il va dans le bon sens et parce qu'il apporte des corrections substantielles, je voterai le texte tel qu'il sera modifié par les amendements du groupe Les Républicains. J'invite tous mes collègues à agir ainsi

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, si nous ne devions retenir qu'un enjeu lié à ce projet de loi, c'est celui de la recherche d'un équilibre entre responsabilité et humanisme, entre répression et laxisme. Cet équilibre est au coeur de l'approche française du fait migratoire depuis trente Ceux qui veulent modifier cet équilibre au profit de l'un ou de l'autre risquent de dénaturer notre modèle d'intégration. Trop de laxisme, d'une part, c'est faillir à l'objectif légitime de lutte contre l'immigration irrégulière. aussi saturer nos services qui font un travail formidable dans des conditions déplorables. C'est enfin se rapprocher des limites de ce que la société française peut intégrer. Trop de répression, d'autre part, c'est méconnaître la tradition française issue des Lumières. C'est se priver de talents qui souhaitent travailler et vivre en France, et c'est risquer de bafouer les droits les plus fondamentaux de la personne humaine. Cet équilibre n'est pas simple à trouver. Il nécessite une approche mesurée. D'un côté, il faut rendre les mesures d'éloignement plus effectives et prendre en compte la dangerosité des candidats à l'asile. De l'autre, il faut accélérer les procédures et moderniser le droit des étrangers. Sur ce dernier point, nous croyons que le droit au travail est un vecteur particulièrement efficace d'intégration et nous vous proposerons des amendements pour en faire une réalité concrète.

Seule une approche structurelle de la question migratoire nous permettra de répondre à la crise que nous connaissons ! La parole est à

souhaite que la protection de l'enfance bénéficie à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les mineurs eux-mêmes. C'est cette approche en faveur de la protection de l'enfant qui justifie que ce sujet complexe et délicat des mineurs non accompagnés n'ait pas vocation à être abordé dans le cadre de ce texte. En la matière, nous espérons que l'État et l'Assemblée des départements de France pourront se mettre d'accord rapidement. Je crois que tel sera le cas, si mes informations sont bonnes.

La démarche que nous négocions avec ces pays repose sur un équilibre entre des incitations négatives, c'est-à-dire des restrictions de visas, comme les projets de coopération. En réalité, nous mettons en équilibre les visas et les laissez-passer consulaires. Nous avons d'ailleurs renforcé le pilotage des demandes et du suivi de la délivrance des laissez-passer consulaires

direction centrale de la police aux frontières. Son rôle consiste à harmoniser les procédures de saisine des consulats par nos préfectures et à appuyer ces dernières dans leurs démarches. Nous avons déjà passé des accords avec le Maroc, la Tunisie, la Guinée, le Mali, la Côte-d'Ivoire et le Sénégal. Les résultats de cette mobilisation sont déjà perceptibles pour plusieurs pays, en particulier après que nous avons utilisé le dispositif de restriction des visas ou lorsqu'un accord de réadmission a été conclu

Cet article, introduit en commission, est tout un symbole. Nous devrions entamer un tel texte par la proclamation de grands principes censés définir notre politique d'accueil et de gestion des migrations, et voilà un article qui, d'emblée, s'attache à un seul objectif : définir pour les

et le seuil à partir duquel sera déclenchée, quoi qu'il en coûte, et quelle que soit la situation, la machine à expulser, à renvoyer et à ignorer les vies ainsi brisées ! Nous sommes là au coeur du problème projet de loi se refusent à regarder en face l'un des enjeux majeurs de l'histoire de l'humanité, celui des migrations. Cet enjeu est partie intégrante de la construction de notre nation nation et prend une importance décuplée, à l'heure de la mondialisation, des dérèglements climatiques et de l'explosion des inégalités. Les humains ont toujours migré pour vivre ou survivre, pour fuir les conditions de vie indignes, pour en chercher de meilleures. Ils migrent aussi pour fuir les persécutions religieuses ou politiques, les guerres, les génocides. Le rapport statistique annuel de l'Agence des Nations unies estime à 65 millions le nombre de personnes déracinées à travers le monde à la fin de l'année 2016, du fait de conflits et de persécutions, la plupart de ces migrations se faisant d'ailleurs du Sud vers le Sud.

4 200 personnes ont été relocalisées en France à ce jour au titre du mécanisme de relocalisation adopté par le Conseil de l'Union européenne.

Après 1915, fuyant le génocide perpétré par l'État turc, 200 000 Arméniens ont été accueillis par notre pays. Nombre d'entre eux furent aussi de ceux qui défendirent la liberté de la France et tombèrent pour elle. À la suite d'un accord entre les gouvernements français et polonais, plus de 700 000 Polonais sont venus apporter leurs bras à une industrie française qui en manquait terriblement. Chassés par le fascisme, 600 000 Espagnols, défenseurs de la deuxième république espagnole, que nous avons abandonnée, ont traversé les Pyrénées durant l'hiver de 1939 pour trouver refuge en France. Je pourrais aussi évoquer les Belges, les Italiens, les Portugais, les Algériens, toutes ces populations qui ont contribué à faire de notre pays ce qu'il est aujourd'hui : une République de citoyennes et de citoyens unis dans la démocratie par les règles communes qu'ils se sont données. Je passe sous silence les migrations passées, comme celles qu'évoque le décor de la salle des conférences avec les Germains de sainte Geneviève et de Clovis, ou celles qui ont fait presque totalement disparaître les premiers habitants des îles des Antilles, ainsi tous les échanges récents qui font que, aujourd'hui, un Français sur quatre a un parent d'origine étrangère. L'identité de la France n'est à chercher ni dans un roman des origines ni dans un discours historique national qui exclut, mais dans cette dynamique perpétuelle qui mêle les populations et les unit dans la défense de valeurs républicaines qui les dépassent. Le philosophe allemand Hegel explique très bien comment, dès qu'une chose est figée, elle est morte et remplacée par autre chose. Ce qui compte le plus dans notre République n'est pas d'où nous venons, mais où nous souhaitons aller ensemble. L'historien italien Massimo Montanari dit l'identité n'existe pas à l'origine, mais au terme du parcours ». Ma conscience républicaine est blessée quand vous présentez, comme vous le faites avec ce texte, l'immigration comme un mal dont il faudrait se prémunir, une maladie qu'il serait nécessaire de réduire et d'endiguer. Je suis triste pour celles et ceux qui, venus d'ailleurs, ont tant apporté à la France, quand je lis qu'il faudrait définir une politique nationale d'immigration et d'intégration « conforme à l'intérêt national L'intérêt de la Nation est justement dans cette recomposition permanente du corps civique, dans cet amalgame infini des différentes cultures !

: « Une politique de contingents migratoires limitatifs serait sans utilité réelle en matière d'immigration de travail, inefficace contre l'immigration irrégulière et, s'agissant des autres flux, incompatible avec nos principes constitutionnels et nos engagements européens et internationaux. » Voilà ce que disait M. Mazeaud il y a dix ans. En réalité, il suffit de réfléchir deux minutes

Karam, sur l'article. Vous m'excuserez de prendre la parole sur l'article, mais je souhaitais insister sur un point avant que nous n'examinions le texte dans le détail. Les flux migratoires exceptionnels

Il est plus que temps de prendre en compte les pressions migratoires extraordinaires qui s'exercent depuis de nombreuses années en Guyane, qui, je le rappelle, est en Amérique du Sud, et à Mayotte, qui, je le rappelle également, est dans l'océan Indien, poussant le système d'accueil et d'intégration au bord de l'asphyxie. Ce système est impossible à gérer aujourd'hui. Voilà quelques mois, lors de l'examen du projet de loi de finances, j'avais alerté notre assemblée sur l'ampleur du phénomène en Guyane en rappelant quelques chiffres. En trois ans, 11 000 demandes d'asile ont été enregistrées par l'OFPRA. Je le répète pour mieux le souligner : 11 000 demandes en trois ans en Guyane, c'est comme si la France comptabilisait chaque année près d'un million de demandes d'asile sur son seul territoire hexagonal. Parce que seuls de tels chiffres nous permettent de prendre la mesure des événements, nous proposerons que le rapport prévu par cet article 1 A intègre une information exhaustive sur la politique d'immigration et d'intégration outre-mer. Vous le savez, ce texte prévoit par ailleurs un certain nombre de dispositions spécifiques à Mayotte et à la Guyane. Pour cette dernière, un décret spécial vise également à expérimenter un traitement accéléré des dossiers. Aussi, tout au long de notre débat, je m'efforcerai de partager avec vous une image juste et mesurée de nos réalités. Si l'asile est un droit qu'il ne faut pas remettre en question, il est aussi un bien précieux que nous devons protéger lorsque celui-ci est dévoyé. Par exemple, il y a moins d'une semaine, en Guyane, un réseau lié à la République Dominicaine a été démantelé à Cayenne, avec l'interpellation d'une personne dont les coordonnées ressortaient dans 118 demandes d'asile ou titres de séjour.

accélérer ne veut pas dire négliger. Il me semble donc indispensable d'améliorer en parallèle les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Guyane. La parole est à M.

que devient l'application de l'article 45 de la Constitution. Nous avions déjà les charmes de l'article 40, les beautés de l'article 41, et, maintenant, voici l'article 45. Aux termes

les foudres de l'article 45 ne s'abattent-elles pas sur cette

Pour des raisons liées aux demandes d'asile, à la misère économique et sociale et aux changements climatiques, les migrations sont appelées à se développer dans les prochaines décennies. La présente législation prend en compte ce mouvement irréversible et vise à y apporter des solutions respectueuses de l'ensemble des êtres humains concernés dans le cadre d'un projet européen qui devra être à la mesure de l'enjeu, et en concertation avec les pays d'origine et les pays d'accueil.

normatives : « Le Parlement détermine pour les trois années à venir le nombre d'étrangers admis à s'installer durablement en France pour chacune des catégories de séjour, à l'exception de l'asile, compte tenu de l'intérêt national. L'objectif en matière d'immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s'attachent à ce droit. »

c'est quand même idiot de demander au Parlement de limiter le nombre de talents étrangers qui voudraient venir en France ; c'est quand même idiot de limiter l'attractivité des universités françaises en laissant le Parlement limiter le nombre d'étudiants venant en France. Je le répète,

Dieu est grand, mais ce n'est pas exactement le problème aujourd'hui. Sincèrement, on ne doit pas vivre dans le même pays ni dans le même monde.

tendant à définir des indicateurs précis de la présence des étrangers dans notre pays. Il s'agit en fait de conforter des improuvés et improuvables dans leur lapidaire expression,

en vertu d'accords de coopération universitaire ? -, c'est que, manifestement, ici, on appelle étrangers tous ceux qui demandent à entrer en France, alors même qu'un grand nombre de ces entrées concernent des Français nés hors de la métropole et, parfois, leurs conjoints et leurs enfants. N'oublions pas que la France pratique en la matière à la fois le droit du sol et le droit du sang. Une étude relativement récente de l'INSEE sur les flux migratoires observés de 2006 à 2013 nous révèle, entre autres informations, que nous avons enregistré pas moins de 2,466 millions d'entrées sur notre territoire, dont 1,633 million d'immigrés, et, de fait, 833 000 Français nés en France ou à l'étranger. Le tiers des entrées sur le territoire national concerne donc des ressortissants hexagonaux. Sur la même période, 2,068 millions de sorties du territoire national ont été constatées, dont plus de 500 000 personnes de nationalité étrangère. Le solde migratoire est passé de 113 000 personnes en positif en 2006 à seulement 33 000 aujourd'hui. De fait, un nombre croissant de jeunes Françaises et Français, faute de trouver un emploi à la mesure de leurs qualifications dans leur propre pays, vont travailler ailleurs, là où l'on sait reconnaître la qualité de la formation scolaire et universitaire hexagonale. Ainsi, on évalue en 2013 à près de 855 000 le nombre de Françaises et de Français âgés de 25 ans à 34 ans résidant à l'étranger, ce qui représente 4 % de notre population active ou plus de 5 % de l'emploi privé.

Les différents éléments mentionnés dans l'amendement voté en commission des lois, dont ceux relatifs à la politique européenne d'immigration et d'intégration, figurent déjà dans ce rapport. Cet article

ne résiste pas à l'examen de faisabilité. Elle n'avait d'ailleurs pas été mise en oeuvre par les gouvernements précédents. Je ne citerai pas Pierre Pierre Mazeaud, puisque M. Yung l'a fait tout à l'heure, mais il avait conclu au caractère irréalisable de ces quotas. Le Gouvernement n'est pas favorable à ce qu'une telle politique soit mise en oeuvre. En effet, l'immigration familiale résulte en grande partie des principes figurant dans la Constitution- le droit à mener une vie familiale normale ou la liberté de mariage -et, bien sûr, dans les conventions internationales. En ce qui concerne l'immigration professionnelle, notre droit encadre l'emploi des nouveaux immigrés par la délivrance des autorisations de travail en fonction de la situation S'agissant des talents internationaux et des étudiants étrangers, dont il a été question à l'instant, le Gouvernement a fait le choix de développer l'attractivité du territoire national pour ces publics, compte tenu de leur apport à notre économie et au rayonnement de la France. les actions conduites par les collectivités territoriales peuvent être déjà ajoutées au rapport en tant que de besoin, sans qu'il soit nécessaire de modifier la loi. Pour toutes ces raisons, il est donc proposé de supprimer cet article.

par la représentation nationale. De surcroît, il est intéressant de connaître les capacités d'accueil que nous pouvons proposer dans le cadre de ces politiques. À cet égard, nous sommes en parfaite coordination avec l'objectif fixé par le texte, à savoir la maîtrise de l'immigration. Sur les chiffres eux-mêmes, la notion de quota peut être assez large ; elle n'est pas forcément absolument rigide. Elle peut porter naturellement sur les titres de séjour, et non pas sur les pays sources. Par ailleurs, s'il est un élément sur lequel nous avons rarement des informations, c'est celui des régularisations.

Au-delà de la position du Gouvernement, que l'on peut comprendre pour des raisons de positionnement global, la vraie question que nous pose cet article 1 A est la suivante : quelles sont les intentions de ceux qui estiment nécessaire de fixer chaque année un quota d'immigration ? Nous avons souligné, dans la discussion générale, que l'effet réel de l'entrée de personnes de nationalité étrangère sur le territoire français était bien moindre que ce que le discours accompagnant cette réalité de notre temps Et nous avons découvert que, sous certains aspects, notre pays était aussi un pays d'émigration, non pas parce que nous aurions une fiscalité insupportable, ce que croient ou tentent de faire croire quelques beaux esprits noyés dans l'idéologie dominante, mais tout simplement parce qu'en l'état actuel des choses, l'économie et les entreprises de notre pays sont parfaitement incapables de tirer parti de l'élévation continue du niveau de formation générale, scientifique et technologique de nos jeunes diplômés, pour en faire le puissant levier de croissance durable qui nous manque. Le problème récurrent que pose la grande appétence des actionnaires de nos entreprises, de la PME au groupe transnational, pour le retour le plus rapide sur investissement sous forme de généreux dividendes n'est sans doute pas

et, de ce fait, des pays francophones. L'immigration n'a jamais été véritablement un phénomène de masse en France, sauf en certaines circonstances exceptionnelles, lorsque la saignée de forces vives causée par un conflit prolongé avait mené à l'arrivée massive de travailleurs étrangers et de leurs familles. Pour ne prendre qu'un exemple, dans un pays comme le Mali, dont la population a quadruplé depuis l'indépendance, qui frise désormais les 20 millions d'habitants, où le fait de partir pour l'étranger est, dans certaines régions, une forme de passage obligé dans l'existence,

il serait interdit au Parlement de se prononcer sur la politique d'immigration, sur la base de critères dont la liste est fixée dans la loi.

révèle l'absence totale de volonté de maîtrise de l'immigration. Il me semble quand même que, compte tenu des possibilités offertes par la France aux personnes qui veulent s'installer chez nous dans des conditions de dignité, il faut maîtriser l'immigration. Eh bien, face à l'absence de maîtrise

de renforcer les droits du Parlement ! Vous noyez le poisson ! Vous savez très bien que, à travers le débat sur cet article, nous abordons la philosophie de notre politique d'immigration et de notre politique d'accueil. Et c'est sur ce point qu'il y a en effet une différence sérieuse entre nous Vous souhaitez une politique extrêmement restrictive, que vous ambitionnez d'encadrer dans des chiffres définis pour trois ans. Pour notre part, nous pensons qu'il faut, au contraire, traiter cette question en prenant la mesure de l'enjeu

Je crains que les quotas, qui sont peut-être de nature à rassurer, ne soient, en réalité, dictés par la peur. Or il faut reconnaître que la peur n'est jamais bonne conseillère. Elle conduit parfois à des renoncements et parfois à des reniements. Je ne voudrais pas faire de procès d'intention, mais la façon dont a été gérée la problématique de l'accueil de l'me paraît avoir été dictée tout simplement par la peur de la réaction de la partie la plus extrémiste de notre population. Cette gestion conduit, d'une certaine façon, à renier la perception

scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Mme Catherine Di Folco. La commission des lois a prévu l'organisation d'un débat annuel sur la politique migratoire et la remise, au préalable, d'un rapport sur la situation des étrangers en France. Le Gouvernement publie déjà un tel rapport, mais il le fait, la plupart du temps, avec un certain retard. Le rapport actuellement disponible a été publié en février 2017 et il porte sur les données de 2015 Le manque de transparence des données relatives à l'asile et à l'immigration est plus que préoccupant. En conséquence, il est proposé d'imposer au Gouvernement de rendre son rapport avant le 1 juin de chaque année. À l'article 33 du projet de loi, l'Assemblée nationale avait prévu la remise d'un rapport avant le 1 octobre, date beaucoup trop tardive pour le prendre en compte lors de la préparation du projet de loi de finances. Les amendements

Or, vous le savez, les outre-mer totalisent à eux seuls plus de la moitié des reconduites à la frontière menées depuis le territoire français. Les chiffres contenus dans le rapport du Gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration sont destinés à éclairer le Parlement et à lui permettre de contrôler que les politiques migratoires conduites sont proportionnées à l'ampleur des entrées illégales dans notre pays. Or, dans les départements de Mayotte et de Guyane, il est évident que la lutte contre l'immigration clandestine menée jusqu'à présent est loin d'être à la hauteur de l'ampleur des entrées irrégulières qui ont lieu quotidiennement dans ces territoires.

Cet amendement vise à inclure dans ce rapport une information exhaustive sur les chiffres de l'outre-mer, spécialement de Mayotte et de la Guyane. Par ailleurs, mais cela fera l'objet de discussions au sujet d'autres amendements, le dernier rapport gouvernemental consacré aux orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration sur les données de l'année 2015. Il me paraît, à ce titre, fondamental de prévoir que ce rapport soit rendu chaque année avant une date qui aura été jugée à la fois réaliste par le Gouvernement et satisfaisante pour la prise en compte de ces données lors de la préparation du projet de loi de finances.

ont largement été occultées par les auteurs de ce projet de loi. C'est la raison pour laquelle, comme mes autres collègues, je souhaite, avec le présent amendement, inciter fortement le Gouvernement à se doter de moyens à estimer le nombre d'étrangers présents dans les territoires d'outre-mer, plus exposés encore à la pression migratoire que le territoire national métropolitain.

un avis défavorable à l'amendement n° 177 rectifié de M. Leconte, qui est un amendement de suppression. Chacun aura bien compris que nous souhaitons ce débat, en tout cas, la commission le souhaite.

La parole est à Mme Catherine Di Folco. Le droit en vigueur prévoit plusieurs motifs de retrait du titre de séjour, notamment lorsque l'étranger a transmis des informations frauduleuses ou a commis l'un des crimes et délits mentionnés à l'article L. 313-5 du code En outre, le déploiement des titres de séjour pluriannuels demande une grande vigilance : lorsque les motifs de délivrance du titre ne sont plus respectés, la préfecture doit le retirer et procéder à l'éloignement de l'intéressé. nous proposons, par cet amendement, que le rapport sur la situation des étrangers en France précise le nombre de titres de séjour retirés par les préfectures, en complément des données sur le nombre de titres de séjour délivrés. Quel

Le Gouvernement et les députés ont souhaité exclure du projet de loi la thématique des mineurs isolés, qui représente pourtant un véritable enjeu, notamment pour les départements. À l'inverse, la commission des lois du Sénat a utilement prévu la création d'un fichier national biométrique des étrangers déclarés majeurs à l'issue de leur évaluation par un département. Dans la continuité du travail de la commission, cet amendement a pour objet d'inclure la thématique des mineurs isolés dans le rapport annuel sur la situation des étrangers en France. Une transparence accrue est indispensable pour mieux traiter cette problématique ! Quel

sur la politique des quotas proposée par la majorité sénatoriale- avec, en première ligne, M. Karoutchi -, nous vous proposons, une dernière fois, de renoncer à une politique

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

l'état du monde et notre responsabilité. Nous vivons un moment où, sur les questions liées à l'immigration,

! Alors, par rapport à ce danger raciste et populiste qui déferle, semble tout submerger et nous rappelle des moments

vivant en France, quelle que soit leur nationalité, y compris par conséquent les Français. Il serait donc contre-productif d'établir ainsi une liste de droits qui relèveraient d'autres domaines que du seul droit des étrangers, et qui pourraient être modifiés dans le futur. Ainsi, les dispositions portant garantie des droits en matière d'hébergement d'urgence ont leur place dans le code de l'action sociale et des familles, et non dans le CESEDA. Le Gouvernement n'étant pas favorable à l'introduction dans un code dédié aux étrangers de dispositions législatives de caractère général concernant d'autres politiques et un public plus large que les étrangers, il émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement. J'estime

dramatique de la situation en Europe. Nous affrontons des problèmes qu'aucun d'entre nous n'aurait imaginés : pour certains pays de notre Europe,

cher collègue, le point de départ de votre raisonnement, de la même manière que nous ne pouvons pas nous satisfaire des fractures qui existent, non pas seulement entre l'Est et l'Ouest, mais aussi entre l'Europe du Sud

à une convergence entre les pays d'Europe, parce que nous ne pouvons pas nous satisfaire de l'éclatement dramatique, que l'on constate aujourd'hui, des risques de repli sur soi et de montée des nationalismes. Nous devons relever un défi collectif

de garder le contact avec les autres pays d'Europe pour parvenir à une forme de dénominateur commun. Certes, l'exercice est d'une particulière complexité, mais c'est toute la responsabilité du Gouvernement.

Il créait deux nouvelles cartes de séjour pluriannuelles, d'une durée de quatre ans, au profit des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides, ainsi que de leurs familles.

lieu, on sécurise le droit au séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire en facilitant leur intégration et leurs démarches administratives. Il est d'ailleurs intéressant de souligner à cet égard,

bénéficiaires de la protection subsidiaire et du statut d'apatride. Sans cette disposition, les frères et soeurs d'un étranger mineur non marié qui auraient bénéficié de la réunification familiale se trouveraient sans titre de séjour à compter de leur majorité. Il convient de régler cette difficulté. D'autre part,

l'accueil de certains demandeurs d'asile, à savoir ceux dont la demande a été admise au titre de la protection subsidiaire. En effet, le droit en vigueur introduit une différenciation de traitement non justifiée entre réfugiés et personnes admises à la protection subsidiaire les premiers obtiennent une carte de séjour pluriannuelle, tandis que les seconds doivent se contenter de cartes annuelles. Cela place les personnes protégées subsidiairement dans une situation d'insécurité juridique importante. Malgré les efforts considérables réalisés par l'OFPRA pour réduire les délais d'examen, il arrive que la durée de protection accordée soit inférieure à la durée totale de la procédure de demande de protection. Mes chers collègues, je souhaite également vous convaincre de la pertinence de cette mesure du point de vue de la régulation de l'activité contentieuse. En effet, le maintien de deux régimes administratifs distincts pose un réel problème.

Sur les autres amendements, je tiens à rappeler que le Gouvernement propose d'octroyer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans aux apatrides et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire dès leur première admission au séjour. Ils bénéficieraient ensuite, au terme de ces quatre ans, d'une carte de résident. Sur ce point, la commission a préféré en rester au droit en vigueur. Le bénéficiaire de la protection subsidiaire recevrait, par exemple, une carte de séjour d'un an, puis une carte pluriannuelle de deux ans. La position de la commission se fonde sur quatre arguments.

Troisièmement, l'article 16 de cette directive prévoit que la protection subsidiaire n'est pas permanente : elle est conditionnée à l'évolution de la situation personnelle des bénéficiaires et, plus largement, des conflits ayant justifié leur protection. En cas de risque permanent, ce n'est pas le statut de protection subsidiaire, mais celui de réfugié, qui doit primer. Enfin, le dispositif proposé par le Gouvernement est moins protecteur pour les apatrides.

à introduire un délai dérogatoire au droit commun pour la délivrance des titres de séjour aux apatrides. Dans l'état actuel du droit, une décision implicite de rejet naît après un délai de quatre mois à compter de l'introduction d'une demande de titre de séjour, quel qu'il soit ; le dispositif proposé dérogerait donc à ce principe. Au-delà, un tel dispositif présente un intérêt limité, puisque la personne concernée reçoit un récépissé, qui est remis dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour et qui permet aux apatrides d'accéder aux mêmes droits que lorsqu'ils sont titulaires de cette carte.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis le début de l'après-midi, nous discutons d'un projet de loi dont le titre sonne comme une incantation immigration maîtrisée », « droit d'asile effectif », « intégration réussie ». Pour autant, le texte proposé par le Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale et remanié par la majorité sénatoriale, durcit le dispositif régissant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers. La Commission nationale consultative des droits de l'homme ne s'y est pas trompée dans son avis sur ce projet de loi, dénonçant son grand danger. En effet, l'esprit est bien loin de la lettre, surtout lorsque ce texte porte sur les populations migratoires les plus fragiles et les plus vulnérables que sont les enfants. Les dispositions s'attachant à la privation de liberté pour ces populations sont choquantes et contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les enfants enfermés ici ou là choquent nos concitoyens. Leur enfermement choque dans le monde entier. Voilà le témoignage du reliquat d'humanité de nos sociétés, de nos civilisations rendues folles par le besoin de réguler les allées et venues des plus faibles

ces derniers obtiendraient ainsi une carte de résident et éviteraient d'être privés du droit de séjour à leur majorité. Il s'agit d'attribuer les mêmes droits à tous les membres d'une cellule familiale et de garantir, conformément à l'article 8

parole est à Mme Michelle Meunier. Il s'agit d'étendre le bénéfice de la carte de résident aux frères et soeurs d'un étranger mineur qui a obtenu le statut de réfugié. En effet, ce projet de loi offre à un mineur isolé

à leur majorité. Faute de quoi, ils se trouveraient sans titre de séjour à leurs 18 ans et seraient donc amenés à devoir quitter la France, alors qu'ils y ont été scolarisés, éduqués et insérés. Quel

aux frères, soeurs, demi-frères et demi-soeurs des mineurs bénéficiant d'une protection internationale. Nous avons bien entendu les arguments de M. Karoutchi ; ils ne convainquent pas : les enfants sont là, on ne va pas les mettre dans des cages, comme font d'autres pays prétendument civilisés ! Il faut donc traiter le problème. Les dispositions actuellement en vigueur sont bien sûr conformes à la directive le droit de l'Union européenne n'interdit pas aux États membres d'adopter des dispositions nationales plus généreuses et contribuant à mieux garantir le droit de mener une vie familiale normale.

Jacqueline Eustache-Brinio. Un mineur devenu majeur est en mesure de déposer une demande d'attribution de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride indépendamment de ses parents. de ses parents. Il s'agit donc de ne plus permettre la réunification que pour les seuls mineurs, en supprimant la phase intermédiaire entre 18 ans et 19 ans durant laquelle de jeunes majeurs peuvent encore rejoindre leurs parents.

a été inscrite dans la législation par la loi relative à réforme de l'asile de 2015. Le Gouvernement souhaite maintenir ces dispositions protectrices, garantes de l'unité familiale et conformes à la directive Qualification. Au-delà, le Gouvernement ne souscrit pas à l'objectif d'exclure les enfants mineurs de la réunification familiale, tandis que les majeurs pourraient y prétendre. Par conséquent, il émet un avis défavorable

n° 34. L'article 3 a trait à la réunification familiale. Il s'agit de l'un des seuls éléments favorables de ce projet de loi qui constituent une avancée concrète pour le droit des réfugiés. Je rappelle que la réunification familiale, qui permet aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides de demander à être rejoints en France par les membres de leur famille, n'est pas le regroupement familial, lequel répond à d'autres logiques, puisqu'il s'applique aux étrangers ne bénéficiant pas d'une protection internationale. Cette procédure spécifique de réunification familiale est fondée sur le principe de « l'unité de la famille reconnu par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par l'article 23 de la directive européenne Qualification du 13 décembre 2011. Initialement, il s'agissait, par cet article, d'élargir le droit à la réunification familiale aux frères, soeurs, demi-frères et demi-soeurs d'un réfugié, d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ou d'un apatride, lorsque celui-ci est un mineur non marié.

Vous avez également argué que les frères et soeurs ont toujours la possibilité « de déposer eux-mêmes une demande d'asile ou de bénéficier d'un visa asile ». Quelle ironie, lorsque l'on sait que l'on parle bien d'enfants mineurs, pour qui ces démarches sont peut-être un peu difficiles à mettre en oeuvre Là où vous évoquez un appel d'air, nous voyons un geste d'humanité. Le fondement même de ce dispositif repose en effet sur les dangers pour la famille restée au pays, notamment les frères et soeurs. Nous demandons donc le rétablissement de cette mesure qui permettra de protéger un certain nombre d'enfants. Très

n° 189 rectifié. Cet amendement a pour objet de rétablir la disposition qui permettra aux mineurs isolés ayant obtenu le statut de réfugié de faire venir leurs frères et soeurs en France. Cette disposition a été supprimée par un amendement au motif que « l'extension du regroupement familial aux frères et soeurs mineurs constituerait un appel d'air pour des flux migratoires toujours plus importants », ce qui illustre à plusieurs titres la confusion entretenue sur ce sujet. D'une part, l'article 3 ne concerne pas le regroupement familial, mais la réunification familiale, laquelle concerne les personnes bénéficiaires d'une protection internationale et leur permet d'être rejoints en France par leur conjoint ou leurs enfants mineurs. D'autre part, en 2016, la réunification familiale a

a dit regretter l'évolution de cet article et la suppression de la réunification familiale. Cet amendement du groupe La République En Marche la rétablit, ce qui est assez logique. Je ne vois pas comment on peut défendre le principe

relatives à la possibilité offerte aux ascendants de mineurs protégés de rejoindre leur enfant au titre de la réunification familiale, en étant accompagnés de leurs autres enfants mineurs non mariés. Il s'agit en effet de préserver l'unité de la famille pour les quelques cas rencontrés chaque année- il n'y en a pas énormément -et l'OFPRA accorde la protection à des mineurs qui bénéficient ensuite du rapprochement familial de leurs parents. Il ne faut pas placer des parents devant le dilemme de devoir rester avec une partie de la fratrie en France ou avec une autre au pays. Certains

En effet, cette disposition concernera peu de monde : en 2017, seuls 357 mineurs ont reçu la protection de l'OFPRA. Ceux qui brandissent la menace d'un appel d'air mélangent volontairement aussi deux phénomènes- je n'accuse personne qui demandent l'asile, lesquels sont peu nombreux- 591 demandes en 2017 -et les mineurs non accompagnés, qui demandent la protection de l'enfance- 54 000 demandes en 2017 adressées aux conseils départementaux. En outre, je tiens à rappeler que la réunification familiale pour les réfugiés est une procédure absolument spécifique et très encadrée. Seules 2 380 personnes sont venues en France à ce titre en 2017. Elle ne doit pas être confondue avec l'ensemble de l'admission au séjour pour les étrangers du fait de la vie privée et familiale, ce que l'on appelle le regroupement familial, mais qui est plus large encore, et dont le chiffre s'élève à 83 478 entrées pour motif familial. Dans ces conditions, le Gouvernement émet bien sûr un avis favorable

sémantique et les métaphores météorologiques convoquées : nous avons eu droit à la submersion, au raz de marée, à l'inondation, au déferlement, au tsunami

et le fait d'employer toujours ces mots a, bien sûr, un effet, et un effet très négatif. De deux choses l'une : ou il y a un droit ou il n'y en a pas. Le droit s'applique à chaque être humain. Nous sommes ici pour essayer de construire le meilleur droit possible.

c'est que l'Europe, dans sa totalité, se dote d'organismes beaucoup plus puissants et de moyens beaucoup plus adaptés, de manière à mettre fin au trafic des passeurs.

Ce dispositif va entraîner une explosion de l'immigration, jetant sur les routes de la mort de nombreux mineurs non accompagnés qui, une fois en France, pourront faire venir légalement non seulement leurs parents, mais également toute leur fratrie.

supposer qu'ils obtiendront satisfaction. Pourquoi est-ce que ce qui nous permettait jusqu'alors d'honorer intégralement notre devoir deviendrait aujourd'hui insuffisant ? la mesure qui a été introduite par l'Assemblée nationale, et que personne ne réclamait, ne présente aucune espèce d'utilité dès lors que ces mineurs étrangers seront reconnus comme réfugiés sans aucun problème.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable

À l'inverse, l'amendement n° 190 rectifié de M. Leconte tend à apprécier l'âge de l'enfant plusieurs mois avant, au moment de la demande d'asile, ce qui conduirait d'ailleurs à admettre à la réunification familiale